vous est donné de votre mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au et figurera dans l'analyse politique du scrutin. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2022

Mayotte. Alors que l'Hexagone compte environ 437 médecins généralistes ou spécialistes pour 100 000 habitants, la Guyane n'en compte que 256 et Mayotte 78, ce qui en fait le plus grand désert médical de France. Le constat du manque d'attractivité des outre-mer est établi, qu'il s'agisse des médecins généralistes ou des spécialistes. Il est ainsi primordial de renforcer l'attractivité médicale de ces territoires particulièrement frappés par la crise sanitaire. Cet amendement vise donc à inciter les médecins nouvellement diplômés à s'installer dans les deux territoires concernés grâce à l'instauration, sous forme d'une expérimentation de trois ans, d'une exonération de cotisations sociales sur les revenus d'activité en cas d'installation dans l'année qui

Cette disposition permet en France à tout journaliste professionnel de collaborer avec un média, d'avoir une sécurité sociale, de travailler dans la sécurité,

un salarié peut bénéficier d'un contrat de détachement s'il en respecte les conditions, c'est-à-dire un travail préalable réalisé en France pour un employeur donné, un lien organique maintenu avec cet employeur et une durée maximale de détachement. Dans ce cas, le travailleur reste rattaché au régime général français et son employeur s'acquitte des cotisations et contributions de droit commun en France.

l'adoption de cet amendement ne modifierait en rien cette dichotomie juridique, issue de règlements européens et d'accords internationaux que la loi ne peut pas ainsi modifier. C'est la raison pour laquelle, même si le sujet nous paraît évidemment intéressant et même si nous sommes prêts à y travailler, l'avis du Gouvernement est, à ce stade, défavorable. La parole est

Nous ne pouvons pas nous contenter de décrire la situation du droit commun d'une personne partant travailler à l'étranger. Cela n'est pas suffisant. Si nous voulons assurer l'indépendance de notre information et des sources,

Ces derniers bénéficient en effet, depuis 2019, de l'abattement de charge pérenne de 8 % de la masse salariale. Il s'agit d'une surcharge d'environ 400 millions d'euros par an du secteur public. Cette différence de traitement pénalise les établissements médico-sociaux publics, qui accueillent la grande majorité des résidents les plus modestes. Il est inéquitable de les surtaxer ou de les taxer différemment par rapport au secteur privé. Les abattements de cotisations sociales doivent donc s'appliquer aux établissements publics. À défaut, ceux-ci se trouvent dans une situation de désavantage concurrentiel, qui pourrait menacer leur pérennité à terme.

et je ne reviendrai pas sur l'épisode « pas de blouse, pas de gel, pas de masque, etc. » Il y a quelques semaines, nous avons examiné la proposition de notre collègue en faveur du droit de visite des patients dans les hôpitaux, dans les centres pour personnes en situation de handicap et surtout en Ehpad. La pandémie a braqué les projecteurs sur un secteur privé à but lucratif, qui cherche à réduire les coûts et à maximiser les les profits. Sur tout le continent européen, des multinationales cotées en Bourse et des fonds d'investissement rachètent des maisons de retraite pour les transformer en machines à cash.

Or le prix de l'hébergement est bien supérieur dans les établissements privés à but lucratif. Ces derniers n'ont donc pas attendu cette taxe pour facturer un prix de journée beaucoup plus élevé.

cliniques privées n'y sont assujettis. Cette taxe ampute chaque année le budget de l'hôpital de 5 milliards d'euros. Le système de tuyauterie entre l'État et la sécurité sociale fait que, chaque année, une partie de cette somme est paradoxalement redéployée vers les différentes branches de la sécurité sociale. C'est pourquoi, une fois de plus, nous appelons à calfeutrer les budgets, car cette taxe revient, en l'état, à mettre à contribution l'hôpital

afin de laisser le temps au Gouvernement de trouver de nouvelles recettes pour le budget de l'État. Et s'il n'a pas d'idées, nous avons des propositions

de l'accompagnement des soins et des services à domicile. Évidemment, des discussions sont en cours sur le partage des charges financières. Sur le principe, cet avenant apporte une véritable revalorisation des emplois, que ce soit en termes de rémunération du personnel

Si les départements sont amenés à amortir cette augmentation sur leurs fonds, il est important de noter qu'il s'agira, pour eux aussi, d'une augmentation significative des dépenses et que tous les départements n'auront pas la même capacité à agir.

et de 50 % pour 2022. Puisque tous les départements ne pourront pas soutenir les services de la même façon, cela entraînera une inégalité de fait entre les différents services d'aides à domicile selon leur département de rattachement.

entre le professionnel ou l'établissement de santé et l'organisme. Il paraît donc cohérent que, dans le cadre de l'action en recouvrement, l'organisme réponde de manière motivée aux intéressés. Tel est l'objet de cet amendement. Quel

Gruny. Cet amendement tend à prévoir la possibilité pour le cotisant qui se trouve en situation de litige sur des cotisations de sécurité sociale de saisir une commission des recours, et non pas de recours amiable, pour se faire entendre. Il s'agit bien ici d'une procédure contentieuse. Il vise aussi à suspendre la procédure en recouvrement des cotisations prévue à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, dès lors que le cotisant conteste la mise en demeure devant la commission des recours.

Pour recevoir l'attestation de vigilance, une entreprise donneuse d'ordres est tenue de vérifier que son cocontractant- l'entreprise sous-traitante -s'acquitte de ses obligations relatives à la déclaration et au paiement des cotisations à l'égard de l'Urssaf. Sans cette vérification, si le sous-traitant a eu recours au travail dissimulé, le donneur d'ordre peut être poursuivi pénalement et devoir régler solidairement les cotisations sociales du sous-traitant. Pour donner à l'entreprise donneuse d'ordres la possibilité de s'expliquer, il convient d'inscrire dans la loi que le refus de délivrance de l'attestation de vigilance ne peut intervenir qu'au terme de la procédure contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou de tout avertissement.

En outre, ce dispositif paraît peu opérationnel, car, en l'absence d'une décision positive, les entreprises concernées ne disposent pas d'une attestation de vigilance.

Mme Pascale Gruny. Concernant la procédure d'analyse de l'activité des professionnels de santé, la loi renvoie à un décret le suivi de la procédure. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce décret n'est pas précis quant au déclenchement de la procédure. Cet amendement vise à ajouter que les intéressés doivent être informés des périodes vérifiées et des pièces demandées, mais également, comme en matière de cotisations dans le cadre de la charte du cotisant contrôlé, de l'existence d'un document intitulé « charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé ». Ce document existe déjà, mais il n'a pas été approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale : il n'est donc pas opposable aux organismes effectuant le contrôle. ? L'avis de la commission était plutôt défavorable, mais je me tourne vers le Gouvernement, parce que nous aurions souhaité des précisions quant à cette charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé et au processus de son approbation. Quel est l'avis

sont déjà portées à la connaissance de ces derniers dès l'engagement du contrôle, puisque les périodes faisant l'objet de la vérification sont couvertes par la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé. Cette charte est systématiquement communiquée dans le courrier adressé au professionnel et l'informant du lancement de l'analyse individuelle d'activité. Il ne nous paraît pas nécessaire d'ajouter cette disposition dans la loi. De plus, mentionner la période contrôlée dès l'envoi de ce courrier n'apporterait rien en termes de droits de la défense, dès lors que cette information est déjà communiquée à l'issue de l'analyse d'activité dans le cadre de la notification des griefs reprochés aux professionnels. Cette notification précède une phase d'échanges contradictoires intervenant elle-même avant l'adoption d'éventuelles sanctions. Je le précise, un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2019 a confirmé l'analyse selon laquelle les modalités d'information du professionnel actuellement prévues par le code sont adéquates pour garantir le respect des droits de la défense. Au bénéfice de ces explications, le Gouvernement sollicite

n° 73 rectifié . Cet amendement a pour objet de placer les entreprises domiennes du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d'exonération de charges sociales patronales spécifique, applicable applicable aux entreprises ultramarines pour une durée d'une année s'étendant du 1 au 31 décembre 2022. Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d'ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86 % de l'activité du secteur.

Mise à mal par ce manque chronique d'activité, la filière réunionnaise du BTP, par exemple, a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d'affaires du secteur a ainsi chuté de 40 % en dix ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de vingt ans. Alors que, dans le contexte sanitaire, les entreprises du BTP ont réussi à maintenir la continuité de l'activité économique, une nouvelle réalité menace la profession. En effet, depuis le début de l'année, nos entreprises du BTP se trouvent confrontées à une flambée des prix des matériaux. Ce phénomène, d'abord observé sur les produits acier, cuivre, bois et PVC, puis sur les autres métaux non ferreux, gagne plus récemment les plastiques, peintures, résines, etc. Il est ainsi courant aujourd'hui de voir des augmentations supérieures à 40 %. à 40 %. En outre, le prix du fret a également beaucoup augmenté pour le transport par containers du fait de la raréfaction des touchers de bateaux dans nos territoires, les armements privilégiant les routes plus rentables compte tenu de la conjoncture mondiale. À cela s'ajoutent également des ruptures d'approvisionnement pour certains des matériaux précités. Compte tenu de son poids dans l'économie et de son importance pour l'activité dans les territoires ultramarins, il est proposé d'alléger le poste coût du travail pour les entreprises du secteur du

En l'état, la réforme mise en oeuvre en 2019 par le Gouvernement ne permet pas de répondre à l'enjeu de la création d'emplois hautement qualifiés dans les outre-mer dans le domaine des TIC et de la recherche et développement. L'amendement

La filière vitivinicole, fleuron de notre économie, enchaîne les malheurs depuis quatre ans- taxe Trump, crise sanitaire qui a fait perdre plus de 1,5 milliard d'euros, aléas climatiques violents, comme cette année le gel généralisé, etc. -à tel point que l'Espagne est passée devant la France cette année en matière de production viticole. Notre économie a donc un genou à terre, et il faudra mettre en place des mesures de très long terme. À court terme, d'ores et déjà, nous souhaitons cet amendement proroger pour l'année 2022 l'exonération des charges sociales pour les exploitants des filières vitivinicoles.

est à Mme Laurence Cohen. Notre collègue Jean-Yves Roux a récemment demandé au Gouvernement de revoir le financement des ruptures conventionnelles pour les petites communes, mais le Gouvernement a refusé d'exonérer ces dernières. Le choix de supprimer les cotisations sociales sur les ruptures conventionnelles dans la fonction publique d'État entraîne non seulement un coût pour la sécurité sociale, mais aussi des inégalités avec les autres secteurs de la fonction publique, notamment la fonction publique territoriale. En abaissant toujours davantage les cotisations sociales, d'un côté, la sécurité sociale est privée de ses recettes, puisque l'État ne compense pas toujours ces exonérations, et, de l'autre, il n'y a pas de renforcement de l'attractivité économique. Au contraire, cela crée un appel d'air, puisque tous les secteurs secteurs demandent le bénéficie des exonérations de cotisations sociales. Ainsi, les exemptions de cotisations du secteur privé ont été étendues à la fonction publique d'État et, désormais, la fonction publique territoriale demande à en bénéficier. Plutôt que d'aligner vers le bas les règles d'assujettissement social sur les ruptures conventionnelles, nous proposons tout simplement de rétablir les cotisations sociales sur l'ensemble des ruptures conventionnelles, et, ainsi, de permettre à la sécurité sociale de dégager de nouvelles recettes pour financer par exemple le développement des crèches dans les collectivités territoriales. Un tel mécanisme est bien plus avantageux que celui du puits sans fond des exonérations de cotisations sociales. sociales. Tel est le sens de notre amendement. L'exonération de CSG prévue dans la limite de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement permet d'aligner le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle sur celui de l'indemnité de licenciement. licenciement. L'assujettissement de l'indemnité de rupture conventionnelle à la CSG rendrait ce mode de rupture de la relation de travail moins avantageux sur le plan indemnitaire que le licenciement.

les plus importantes. Avec la crise sanitaire, nous pensions en avoir terminé avec les parachutes dorés, mais récemment l'affaire d'un ancien président du Crédit Mutuel Arkéa refait parler de ce système fiscal qui interroge à plusieurs niveaux. Par exemple, le code de gouvernement d'entreprises des sociétés cotées de l'Association française des entreprises privées et du Medef, qui prévoit que le versement d'indemnités de départ à un dirigeant mandataire social doit être exclu,

L'ancien président de cette filiale du Crédit Mutuel devrait ainsi toucher 2,5 millions d'euros d'indemnités de rupture. Le contrat de retraite chapeau, qui est souvent présenté comme un outil de fidélisation des cadres supérieurs de l'entreprise, fait l'objet de scandales réguliers dans la presse, avec des rémunérations exorbitantes versées à certains grands patrons. Nous proposons d'augmenter les cotisations sur ces contrats de retraite, en faisant passer le

percevaient une rente annuelle supérieure à 5 000 euros en 2012 et étaient donc redevables de la contribution supplémentaire. Bien qu'une augmentation de la contribution sur la partie supérieure à 24 000 euros par mois ne soit pas inenvisageable par principe,

Le PLFSS pour 2020 a abaissé le taux de cotisations sur les actions gratuites

Ce dispositif d'attribution gratuite d'actions concerne essentiellement des personnes très bien rémunérées de grands groupes et les dirigeants. En plus du coût non négligeable qu'il a pour les finances sociales,

dans les taxations que l'on demande, je n'arrive pas à comprendre que le Gouvernement ne se saisisse pas de ces idées, qui sont bonnes, parce qu'elles permettraient une rentrée supplémentaire de recettes, même en modulant les taux différemment. Je ne comprends pas que la commission des affaires sociales,

sur les actions gratuites voté en 2019. Cette disposition, chiffrée à 120 millions d'euros au moment des débats en séance, n'est pas justifiée, alors que le déficit de la sécurité sociale repart à la hausse en raison de l'épidémie

afin de favoriser la distribution d'actions gratuites aux salariés, j'y insiste, des entreprises. Cette nouvelle modification du taux de la contribution, qui serait la quatrième depuis 2015, nuirait à la fois à la lisibilité et à l'attractivité d'un dispositif permettant d'encourager l'actionnariat salarié. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable

Comme nous avons l'habitude de le faire, nous demandons l'ajout d'un article proposant de majorer de 10 % les cotisations d'assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salariés comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salariés à temps partiel, et ce afin de limiter le recours à cette forme d'emploi. La corrélation entre le temps de travail et le genre est indéniable. Rappelons que, depuis plus de quarante ans, les femmes occupent 80 % des emplois à temps partiel et que la plupart des métiers concernés par ces contrats se situent dans des secteurs d'activité majoritairement féminins. Ils sont de surcroît dévalorisés par de faibles rémunérations. Dans ces secteurs peu protégés, la flexibilisation a entraîné une précarisation des conditions de vie, de plus en plus de travailleurs et de travailleuses à temps partiel étant contraints de cumuler des emplois pour subvenir à leurs besoins. Rappelons également que, depuis le 3 novembre, à 9 heures 22, les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année. En effet, malgré l'inscription dans la loi du principe d'égalité salariale, les femmes gagnent 16,5 % de moins que les hommes, contre 15,5 % l'an passé. Ce chiffre est en hausse constante depuis 2018. Inégalités salariales et temps partiels contraints s'additionnent pour renforcer ces inégalités et fragiliser la situation des travailleuses. Il ne s'agit pas de nier l'aspiration d'une partie de nos concitoyennes et de nos concitoyens à travailler moins et à se libérer du temps pour d'autres activités. Mais pour cela, il suffirait d'abaisser le temps de travail légal. C'est pourquoi nous proposons cet amendement, qui vise à nous rappeler que la sécurité sociale constitue un

la commission ? Nous avons eu l'occasion, voilà quelques jours, de débattre sur l'égalité entre les hommes et les femmes et de défendre un même traitement

en lieu et place de l'année pose question en cas de décès de l'exploitant. En effet, le résultat de cessation d'activité, souvent important eu égard aux caractéristiques des exploitations agricoles, se trouve intégralement soumis aux prélèvements sociaux. Il faut à tout prix éviter que le résultat fiscal de cette cessation d'activité non prévue n'aboutisse à un appel de cotisation trop important. L'option réalisée pour une période minimale de cinq ans révocable annuellement serait ainsi réputée révoquée par l'effet de la loi en cas de décès. De la même façon que la loi prévoit une proratisation des cotisations l'année du décès, un basculement automatique sur la moyenne triennale permettrait d'encadrer le paiement des cotisations sociales dues après le décès de l'exploitant. de la commission ? L'option pour le calcul des cotisations sociales des agriculteurs sur la base des revenus de l'année précédente, au lieu de la moyenne des revenus des trois dernières années, est souscrite pour cinq ans. Cet amendement vise à prévoir que, en cas de décès, cette option serait réputée révoquée, et ce au motif que la moyenne des revenus des trois dernières années constituerait une assiette plus favorable que les revenus de l'année précédente.

la bascule vers une assiette fondée sur la moyenne des revenus des trois dernières années serait moins favorable que le maintien de l'option pour les revenus de l'année précédente. La mesure proposée ne paraît donc pas adaptée à toutes les situations. Méfions-nous : cette

aux agriculteurs de faire face à ces difficultés.

L'assiette sociale doit évoluer, pour donner la possibilité aux agriculteurs de cotiser au plus près de la réalité de leurs derniers revenus. La démarche conduite pour l'impôt avec la mise en oeuvre du prélèvement à la source doit être transposée à l'assiette des cotisations sociales. sociales. Certains exploitants souhaitent bénéficier d'une assiette variant peu d'une année sur l'autre, lorsque d'autres souhaitent une assiette qui soit la plus proche possible de leurs revenus de l'année. Sans remettre en cause l'assiette triennale, qui demeure le régime de droit commun, il est donc proposé de permettre aux agriculteurs, dès 2022, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l'année, en lieu et place de l'option pour

nous rétablirions une véritable égalité entre travailleurs indépendants artisans ou commerçants, qui sont placés sous le régime de la sécurité sociale, et travailleurs indépendants agriculteurs, qui se trouvent sous le régime de la MSA. La parole

vote. Cette situation mérite effectivement d'être prise en considération, notamment dans le vignoble. Avec les aléas climatiques, il y a vraiment des différences de récolte d'une année sur l'autre.

? Cet amendement vise à permettre aux employeurs comme aux travailleurs indépendants des départements et régions d'outre-mer, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon,

en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire. Je rappelle que le décret du 25 mars 2021 fixe la durée maximale d'apurement à trois ans et permet de porter cette durée à cinq ans pour les employeurs et les travailleurs indépendants de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy déjà bénéficiaires d'un plan d'apurement. Il ne semble pas opportun d'étendre cette dérogation prévue à la suite du passage de l'ouragan Irma à des territoires qui n'ont pas été frappés par cet épisode climatique. L'avis de

d'un délai supplémentaire pour rembourser les dettes sociales accumulées à l'occasion de la crise du covid. En réalité, votre demande est plus que satisfaite, puisque j'ai annoncé, à l'occasion du débat à l'Assemblée nationale, que le décret que Mme la rapporteure générale vient de citer et qui fixe à trois ans

Je remercie M. le ministre de sa compréhension- j'allais presque dire de sa générosité. J'avoue n'avoir pas compris les motifs invoqués par Mme la rapporteure

de revenir sur la négociation de la convention d'objectifs et de gestion 2021-2025 entre l'État et la MSA (COG 2021-2025). Le 26 mai dernier, devant la commission des affaires sociales du Sénat, le président et le directeur agricole (CCMSA) ont tiré la sonnette d'alarme sur la situation de la MSA et les conséquences des efforts de mutualisation du réseau avec d'autres régimes. Je rappelle que cet organisme a déjà perdu 4 000 emplois temps plein travaillés en dix ans. La COG 2021-2025 demande d'en supprimer encore 1 500. Ces baisses d'effectifs, associées à la réduction de 5 % des charges de fonctionnement, font craindre, à terme, la disparition du régime agricole. Je mets aux voix

qui précomptent les cotisations et contributions sociales des artistes-auteurs auxquels ils versent une rémunération sont dans l'obligation de remettre à ces derniers un certificat de précompte

L'article 13 prévoit, pour pallier ces défaillances, que l'Urssaf met à la disposition des artistes le certificat de précompte correspondant aux cotisations et contributions sociales reversées par les EPO. Il paraît toutefois nécessaire d'améliorer la qualité rédactionnelle de cet article, afin, d'une part, de garantir que ce certificat porte bien sur l'ensemble des cotisations et contributions sociales dues par les artistes-auteurs, et, d'autre part, d'éviter toute confusion entre cette nouvelle obligation pesant sur l'Urssaf

sur ce sujet, en votant cette année la revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles pour les femmes, les conjoints collaborateurs et les aides familiaux. Il convient d'aller plus loin en sécurisant davantage ces statuts et en limitant les trappes aux basses retraites,

limitation de cinq ans, à la condition qu'elles cotisent, à l'expiration de ce délai, sur une assiette au moins égale à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale,

: la création de cette formule visait précisément à reconnaître l'activité non rémunérée de conjoints contribuant à la gestion de l'entreprise, de façon à leur permettre de disposer d'un statut et d'une couverture sociale.

de ses droits sociaux, notamment au titre de l'assurance vieillesse, tout en maintenant cette liberté de choix entre les trois statuts de conjoint associé, conjoint salarié et conjoint collaborateur.

et à M. le ministre que, décidément, chaque fois qu'il est question des conjoints collaborateurs, c'est-à-dire de femmes dans 99,9 % des cas, on nous rappelle toujours au principe de réalité.

Le présent amendement vise, dans ce cadre, à permettre aux conjoints de chefs d'entreprise ayant le statut de conjoint collaborateur de conserver ce statut sans limitation de durée si, dans le même temps, ils sont travailleurs indépendants à l'extérieur ou salariés dans une autre entreprise.

-que, depuis le 1 novembre dernier, ces retraites ne peuvent être inférieures à 85 % du SMIC. André Chassaigne, avec la constance et la détermination qu'on lui connaît,

Alors que notre pays compte 3,6 millions de chômeurs sans activité, la réduction du temps de travail de 35 heures à 32 heures permettrait de donner du travail à 2 millions de personnes privées d'emploi.

dès 1999. De la même manière, l'usine Bosch de Vénissieux applique les 32 heures à ses salariés depuis 1998 ; elle a réalisé une centaine d'embauches. Cette proposition n'est donc ni illusoire ni impossible à mettre en oeuvre. La crise sanitaire a conduit à la suppression de centaines de milliers d'emplois. Il paraît donc urgent de mieux répartir le temps de travail, en réduisant le temps hebdomadaire travaillé par

sur l'article. Monsieur le ministre, plutôt que de demander un rapport qui sera refusé, je souhaite vous alerter sur le phénomène désormais assez répandu des installations et désinstallations de médecins. En effet, comme vous le savez, dans les zones de revitalisation rurale, les médecins qui créent ou reprennent un cabinet médical peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'un régime fiscal avantageux pendant près de huit ans : une exonération totale d'impôt sur les bénéfices pendant cinq ans, suivie d'une exonération partielle pendant les trois années suivantes.

lui permettant de bénéficier une nouvelle fois de ce régime fiscal, sous réserve qu'il ne reprenne aucun de ces moyens d'exploitation antérieurs et qu'il ne transfère pas sa patientèle. Ce régime induit en fait un effet de bord- une forme de nomadisme médical que l'on constate parfois. C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande de vous pencher, si ce n'est déjà fait, sur ce sujet, à savoir mesurer le nombre de médecins qui bénéficient de cette exonération et, parmi ces derniers, le nombre de médecins qui quittent le département à l'issue de cinq ou huit ans, le nombre de médecins qui bénéficient plusieurs fois de l'exonération fiscale et le coût financier de cette disposition dans son aspect répétitif. Enfin, pour rattacher mon intervention au titre du chapitre III de ce projet de loi, « Poursuivre les actions de lutte contre la fraude », je rappelle que cette disposition extrêmement avantageuse n'est pas un dû, qu'elle n'est pas renouvelable indéfiniment, qu'elle doit être l'objet de contrôles, qu'elle est assortie de conditions- les services fiscaux y sont-ils suffisamment attentifs ? -et qu'elle est discriminante pour les praticiens qui sont fidèles à leur territoire et pénalisante pour les patients. L'amendement

d'obtenir le choix du support de transmission des informations, en l'occurrence d'exiger des documents par voie dématérialisée. Si je ne doute pas que cela puisse faciliter le travail des agents chargés des contrôles- on sait combien le manque d'effectifs est, là aussi, criant ce que je dénonce, avec mon groupe, c'est bien l'entrain général à tout mettre en oeuvre pour effectuer ces contrôles. C'est d'autant plus flagrant qu'une certaine passivité, pour ne pas dire une absence totale de volontarisme, existe à l'égard de la fraude patronale.

La Cour des comptes reconnaissait elle-même la difficulté à évaluer cette fraude. Néanmoins, si nous ne cautionnons pas les fraudeurs, nous dénonçons une nouvelle fois la chasse et la stigmatisation qui se cachent mal derrière cette volonté de lutter contre la fraude aux prestations sociales. De plus, les sanctions contenues dans cet article- entre 1 500 euros et 5 000 euros -nous semblent disproportionnées. Quand il y aura le même allant à lutter contre la fraude patronale et contre l'évasion fiscale qui plombe notre système de protection sociale, notre appréciation différera peut-être. En attendant, nous demandons la suppression de l'article 15. Quel

aux organismes de recouvrement la capacité d'avoir les mêmes facultés que celles qui sont déjà données à l'administration fiscale et à Pôle emploi.

Imbert. Il se revendique comme une série de mises en cohérence sur les contributions des produits de santé. L'un des enjeux est bien d'assurer la bonne intégration de dispositifs dérogatoires de prises en charge dans les différentes assiettes de contribution, particulièrement dans celle de la fameuse clause de sauvegarde, que j'ai essayé d'apprivoiser. Sur le fond, la commission a pu partager, en partie au moins, cette intention et a validé une partie du dispositif. Toutefois, un nombre important de questions se sont posées lors de l'examen de cet article.

sauvegarde : le montant M pour le médicament et le montant Z pour le dispositif médical sont des montants, et non des taux, au-delà desquels les industriels sont redevables de contributions très fortes.

Loin d'un saupoudrage, il faut que nous puissions avoir une position sérieuse et crédible. La commission s'y est attachée. Sur ce point, je regrette d'avoir à constater que la transparence sur la construction de ces montants nous donne malheureusement peu de marge de manoeuvre.

évoquer la situation de la recherche pharmaceutique et le nouveau dispositif d'accès direct des médicaments innovants. La France investit 2,2 % du PIB dans la recherche publique et privée, ce qui la place sous la moyenne des pays de l'OCDE, qui est de 2,4 %. Depuis 2000, le désinvestissement dans la recherche a entraîné une dégradation des conditions de travail des chercheurs. Il me semble que c'est l'occasion ici de réaffirmer qu'il serait

: quand les entreprises licencient, cela a des conséquences économiques et sociales. Notre pays dispose pourtant d'atouts importants en matière de recherche avec l'Agence nationale de la recherche, l'Institut national ; ces trois structures ont connu elles aussi une réduction très forte de leur budget de recherche et le départ de nombreux chercheurs vers la recherche privée. Cette dégradation s'est ressentie lors de la pandémie, avec des retards de certains industriels pharmaceutiques pour trouver un vaccin contre la covid-19. À l'occasion d'un Conseil stratégique des industries de santé (CSIS), le Président de la République avait pourtant annoncé l'accélération de la procédure de commercialisation des médicaments innovants. C'est un autre sujet, mais cette nouvelle procédure pose la question de l'équilibre entre sécurité sanitaire et accès aux traitements innovants. On peut s'interroger sur la pertinence d'accélérer encore les procédures de mise sur le marché des médicaments au regard des scandales sanitaires

qui aide en priorité les fabricants de génériques, dont les remises sont d'ailleurs les plus importantes, avec un plafond à 40 %. Toutefois, si elle me semble pertinente, cette mise en cohérence

donc de les exclure de la clause de sauvegarde.

en matière d'approvisionnement de médicaments. Face à cette situation, il est indispensable de relocaliser en Europe la production, le conditionnement et la distribution des médicaments, nous en sommes tous d'accord. de septembre 2020, la Ligue contre le cancer a publié une étude dressant un constat alarmant en oncologie, puisque trois quarts des professionnels de santé sont confrontés à la problématique des ruptures de stock, et 70 % des oncologues confrontés à ces pénuries de médicaments contre le cancer considèrent que celles-ci auront un impact sur la vie à cinq ans de leurs patients. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 consacre l'obligation pour les industriels de constituer, pour chaque médicament, un stock de sécurité de quatre mois. Or le décret du 30 mars 2021 a révisé à la baisse cette obligation à deux mois

ce sujet ayant été déclarés irrecevables, cet amendement vise à apporter une solution à l'objectif de souveraineté sanitaire et à la lutte contre les pénuries de médicaments. Cette proposition nous paraît plus efficiente que la possibilité de prendre en compte le principe de la sécurité d'approvisionnement du marché français

Loin de moi l'idée de ne pas être sensible à leur devenir, mais je rappelle tout de même que les entreprises pharmaceutiques se portent vraiment très bien. Ainsi, directeur de Sanofi, Paul Hudson, touche un salaire annuel d'environ 12 millions d'euros ; il est le troisième patron le mieux payé du CAC 40. Le bénéfice net de ce grand laboratoire a connu une hausse de 340 % en 2020, passant à 12,3 milliards d'euros. Les dividendes ont connu leur vingt-septième année consécutive de hausse, s'élevant à plus de 4 milliards d'euros. Pourtant, malgré ces profits vertigineux, Sanofi, qui a été incapable de sortir un vaccin contre la covid-19, annonce encore cette année 1 700 licenciements, dont plus de 1 000 en France. Aussi est-ce bien le moins que de demander d'être plus exigeant sur la contribution de ces entreprises en cas d'évolution aussi massive de leur chiffre d'affaires. C'est pourquoi nous proposons de réévaluer à la baisse, et non à la hausse, comme le prévoit l'article 16, les montants Z et M.

l'ensemble des dépenses, quel que soit le type de médicaments. Je rappelle également que la loi de financement de sécurité de la sécurité sociale pour 2019, qui mettait en oeuvre les engagements du CSIS 2018 a justement amélioré amélioré la lisibilité de la régulation macroéconomique des médicaments en intégrant l'ensemble des médicaments dans l'assiette de la taxe, et ce sans exception. Elle a permis d'accroître

sauvegarde. Je précise par ailleurs que les contributions au titre de cette clause ne pèsent pas de la même manière sur l'ensemble des laboratoires, puisque le calcul de la contribution due est fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Elles pèsent donc proportionnellement moins sur les laboratoires dont les produits sont les moins coûteux, comme les exploitants de génériques ou de biosimilaires.

L'amendement n° 827 a pour objet d'abaisser le montant de la clause de sauvegarde des médicaments et des dispositifs médicaux. Nous partageons évidemment cette volonté de réguler efficacement les dépenses associées aux produits de santé, ce qui est indispensable pour assurer la soutenabilité de notre système. Pour autant, l'objectif des clauses de sauvegarde est de contenir la progression de la dépense, laquelle est liée, certes, à une hausse des coûts de traitement, mais également à un vieillissement de la population et à l'arrivée en miroir d'innovations thérapeutiques au fil des années. Par conséquent, abaisser les niveaux des clauses de sauvegarde par rapport à l'année précédente, comme tend à le prévoir cet amendement, irait à l'encontre des industries de santé (CSIS) du mois de juin dernier, qui annonçait une croissance de 2,4 % en moyenne sur la dépense remboursée des produits de santé pour la période 2022-2024, justement pour permettre d'accueillir l'innovation en France et de pouvoir répondre à des besoins nouveaux

En omettant de prendre en considération le niveau de croissance des entreprises, les modalités actuelles font peser une charge financière additionnelle injustifiée sur les exploitants qui n'auraient pas participé à la croissance du marché. Cet amendement vise à rétablir une règle de calcul équitable et adaptée pour la répartition du montant à payer de la clause de sauvegarde et à permettre ainsi une juste régulation et une juste répartition entre laboratoires.

pour apporter plus de prévisibilité, notamment pour les entreprises, et davantage de cohérence entre le mécanisme et son objectif de régulation. La répartition de la contribution entre entreprises est depuis lors fondée uniquement sur le chiffre d'affaires, et non plus sur le système hybride qui existait auparavant et qui mêlait

est à M. Alain Milon. Concernant les dispositifs médicaux, l'article 16 prévoit l'élargissement de la clause de sauvegarde aux dépenses liées au dispositif de prise en charge transitoire des dispositifs médicaux, plus connu Cette disposition semble particulièrement contestable dans la mesure où elle revient à faire financer, lorsque la clause se déclenche, au moins en partie, les produits très innovants issus du dispositif d'accès précoce par les entreprises elles-mêmes. En outre, il s'agit d'innovations financées par le biais d'un processus dérogatoire. Cette mesure apparaîtrait comme désincitative pour les entreprises aspirant au dispositif d'accès précoce. Or, avec un taux d'évolution du taux Z comparable à ceux des dernières années, cette extension de l'assiette de la clause ne peut que contribuer, précisément, à augmenter le risque de son déclenchement, alors que la clause de sauvegarde est régulièrement présentée,

dans ces hypothèses de construction des montants M et Z. On sait que, sur le montant M, les entreprises sont assez satisfaites des choix qui ont été faits. Pour celles qui produisent des dispositifs médicaux, la définition varie

rapporteure générale. Certaines contributions sont, de par leur construction même, fragiles. C'est le cas de la clause de sauvegarde du dispositif médical. Si différents sujets méritent d'être soulevés et ajustés sur la construction de cette contribution, nous avons voulu de nouveau insister sur son caractère infondé. En effet, en cas de dépassement du montant Z, cette contribution emporte l'intégralité du dépassement. Un taux de 100 % dès le premier euro de dépassement ne me semble pas cohérent. Le présent amendement vise ainsi, sur le modèle de la clause de sauvegarde du médicament, à prévoir un barème progressif en cas de déclenchement de la clause de sauvegarde. Je pense par ailleurs qu'une réflexion doit s'ouvrir pour procéder à d'autres ajustements sur cette clause de sauvegarde, qui, on le voit, a été conçue rapidement et n'est pas aboutie. Elle doit mieux prendre en compte les remises que peuvent consentir les industriels, alors que le mécanisme de déclenchement n'incite pas nécessairement à ces remises. Surtout, nous devons l'avoir à l'esprit, ce secteur du dispositif médical est extrêmement hétérogène, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, avec de grandes entreprises très innovantes, au chiffre d'affaires dynamique,

elles ne sont pas sur les mêmes créneaux de dispositifs médicaux. Ces réalités doivent se retrouver dans un mécanisme fiscal inévitablement commun à l'ensemble du secteur. C'est ce que nous appelons de nos voeux. Quel est l'avis

Comme les années précédentes, le Gouvernement émettra un avis défavorable. Vous dressez de nouveau une analogie avec le médicament, je rappelle que la clause de sauvegarde Z pour les dispositifs médicaux ne concerne que l'hôpital, qu'elle porte sur les montants remboursés et non sur les chiffres d'affaires, qu'elle vise un champ restreint, contrairement aux médicaments qui portent eux sur une base très large, et qu'elle ne s'est pas déclenchée pas depuis son instauration.

L'article 16 ajoute dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments les dépenses afférentes aux médicaments pris en charge au titre d'un accès précoce. Cet amendement vise à préciser que les médicaments

l'AMM, les médicaments ne peuvent faire l'objet d'une publicité auprès du public et des professionnels de santé. La contribution ne pèsera donc pas pour ces médicaments : tout médicament sans dépenses de promotion associées ne fera pas l'objet d'un appel de cette contribution, sans qu'il soit nécessaire de les exclure expressément de son champ d'application. Ensuite, votre amendement tend

parole est à Mme la rapporteure générale. Les contributions sur les produits de santé souffrent d'assiettes dissociées et incohérentes entre elles, parfois dans leur principe même. La commission a souhaité apporter une mise en cohérence supplémentaire pour ce qui concerne la taxe sur le chiffre d'affaires. En effet, les remises consenties par les entreprises demeurent comptées comme du chiffre d'affaires réalisé, ce qui, sur le fond, est contradictoire avec la notion même de remise et avec les efforts consentis sur les prix. Le présent amendement vise donc à prévoir la déduction de ces remises de l'assiette retenue pour la contribution sur le chiffre d'affaires.

Ces remises sont conclues dans le cadre de conventions signées entre les laboratoires et le comité économique des produits de santé, prévues par la loi. Elles permettent de fixer le prix de vente des spécialités pharmaceutiques, puisque celui-ci prend en compte les éventuelles remises que le laboratoire sera contraint de verser en cas de dépassement des volumes de ventes également prévues par la convention. J'ai bien dit « contraint », car, en réalité, ces remises sont non pas des remises consenties, comme le seraient des remises commerciales accordées par les laboratoires à leurs clients, mais bien des sanctions contractuelles, au sens juridique du terme, acceptées par le laboratoire, mais dont le mécanisme est prévu par la loi. C'est l'ensemble du système qui est construit ainsi. Par ailleurs, ces remises permettent aux laboratoires, lorsqu'ils doivent effectivement les payer, d'être dispensés pour tout ou partie de participation à la clause de sauvegarde, ce qui est bien normal, puisque la loi les a créées notamment à cet effet. Pour conclure, ce changement d'assiette modifierait de manière significative les paramètres de la contribution et amoindrirait les recettes perçues par l'assurance maladie

M. Martin Lévrier. Les médicaments dérivés du sang font partie des spécialités exclues de l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires versée par les entreprises pharmaceutiques au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), tout comme certains médicaments génériques et orphelins. Ces médicaments, destinés au traitement de maladies rares et graves, sont essentiels. C'est pourquoi le choix a été fait de les exonérer, afin que l'approvisionnement du marché français ne soit pas perturbé.

Ainsi, une grande partie des médicaments dérivés du sang disponibles sur le marché français est assujettie à cette contribution. Dans ce contexte, le présent amendement vise à exonérer l'ensemble des médicaments dérivés du sang de la contribution sur le chiffre d'affaires qui est versée par les entreprises pharmaceutiques au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

tension, structurelle, du fait de la croissance de la demande mondiale, mais aussi nationale, et conjoncturelle, du fait de la baisse de la collecte de plasma à l'échelle mondiale pendant la crise sanitaire. Dans un contexte de tensions et pour garantir un arsenal thérapeutique le plus large possible, la France a recours à des médicaments dérivés du sang

Par ailleurs, des travaux sont en cours avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les laboratoires qui font appel aux dons rémunérés, pour trouver des réponses structurelles pour l'approvisionnement des patients français. français. Ces travaux ne doivent toutefois pas conduire à fragiliser le modèle éthique français, auquel nous sommes tous très attachés, qui revêt par ailleurs un caractère très sensible pour les associations de donneurs, fournisseurs de matières premières pour les associations de malades. des travaux qui sont en cours, des efforts de financement qui sont déjà réalisés par ailleurs pour améliorer l'attractivité du marché national et du besoin de protéger notre modèle français, je vous suggère donc de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, nous y serions défavorables.

plus particulièrement le cas encore pendant la crise sanitaire, ce dont je veux les remercier. Il est vrai qu'ils exercent une mission de service public, mais, en l'occurrence, ils ont fait le maximum pendant cette crise de la chaîne de dispensation.

mais sur des manquements graves et caractérisés, commis notamment par ces professionnels que je considère comme quelque peu hors la loi. Cet amendement vise ainsi à bien caractériser la récidive et le comportement des par la par la notion de « manquement grave et répété constituant un risque pour la sécurité d'approvisionnement ». Je pense que nous répondons ainsi à la préoccupation de nos collègues. Quel est

de ne pas toucher au terme de « récidive », qui, certes, recouvre des situations très diverses, mais que les autorités chargées de sanctionner les entreprises coupables savent parfaitement analyser

Les publicités pour les paris sportifs, notamment, font l'objet de campagnes publicitaires intenses pendant les compétitions de football, comme cela a été constaté en 2021 pendant l'Euro de football. Ces publicités ont été largement critiquées par les médias et l'opinion publique, car elles incitent fortement à des pratiques de jeu excessives. Aujourd'hui, quelque 40 % du chiffre d'affaires des opérateurs de jeux d'argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive du jeu, et les jeunes sont six fois plus susceptibles d'adopter un comportement problématique. En s'acquittant d'une taxe allouée à la sécurité sociale, les opérateurs de jeu contribuent à diminuer les risques addictifs inhérents à leur secteur d'activité. Par ailleurs, les sommes issues de la taxe permettront de renforcer les missions de contrôle et de prévention du jeu

Tournés majoritairement vers les plus jeunes, ces jeux en ligne peuvent en effet provoquer une addiction élevée chez les plus fragiles, avec des conséquences sociales et sanitaires graves. C'est ce que pointe l'Autorité nationale des jeux, qui dénonce les stratégies de marketing, avec un ciblage renforcé auprès des plus jeunes, et souligne que trois parieurs en ligne sur quatre ont moins de 34 ans.

cette addiction, je l'ai dit, peut avoir des impacts sociaux graves, car elle touche majoritairement une population plus précaire. Selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), les pratiques à risque modéré ou excessif se rencontrent chez des hommes plus jeunes, issus de milieux sociaux modestes, ayant un niveau d'éducation et des revenus inférieurs à ceux des autres joueurs. pratiques se montrent aussi particulièrement dangereuses sur le plan sanitaire. Le jeu d'argent est effectivement l'une des addictions les plus suicidogènes : le nombre de tentatives de suicide est quinze fois supérieur à celui de la population normale.

sportifs en ligne apparaît désormais comme un impératif social et sanitaire. D'où cet amendement, dont l'objet est de limiter la publicité en ligne afin de réduire l'exposition des plus jeunes, en taxant les investissements publicitaires des opérateurs et en reversant les bénéfices de cette taxe à la branche maladie de la sécurité sociale.

de prévention et de santé publique, nous proposons de mettre à contribution les messages publicitaires portant sur les jeux en ligne et paris sportifs. Entre 2014 et 2019, les investissements publicitaires des opérateurs de jeux en ligne et de paris sportifs ont augmenté de 25 %. Ils donnent lieu à des campagnes publicitaires intenses et particulièrement ciblées sur les jeunes D'après les chiffres de la nouvelle autorité de régulation, l'Autorité nationale des jeux (ANJ), trois parieurs en ligne sur quatre ont moins de 34 ans, et l'on sait combien ce public est particulièrement vulnérable aux phénomènes d'addiction. L'un des principaux centres de soins dédiés à Paris, l'hôpital Marmottan, a observé que les jeunes adultes de moins de 25 ans représentaient, à eux seuls, 62 % de la totalité des patients pris en charge pour leur addiction aux paris sportifs. En 2019, l'OFDT relevait dans une étude que les pratiques de jeu à risque modéré ou excessif se rencontrent chez les hommes plus jeunes, issus de milieux modestes, ayant un niveau d'éducation et des revenus inférieurs à ceux des autres joueurs. Grâce au travail de l'ancien Observatoire des jeux- je tiens ici à saluer l'implication de Jean-Michel Costes, qui fut le premier, dès 2011, à nous alerter sur les dangers de ce phénomène -, il est désormais admis que cette pratique peut entraîner de graves troubles de graves troubles sanitaires et psychiatriques et qu'il y a là un véritable enjeu de santé publique. Le présent amendement vise donc à limiter la publicité en ligne, afin de réduire l'exposition des plus jeunes, en taxant les investissements publicitaires des opérateurs. Je précise que le marché du jeu en ligne et de hasard représente plus de 48 milliards d'euros de mises. La parole

jeux. Le présent amendement pourrait être un premier pas vers la prévention des risques liés aux pratiques excessives du jeu, qui touchent les personnes les plus vulnérables, grâce à l'instauration d'une taxe sur les publicités relatives aux jeux d'argent en ligne.

inscrits aux articles 302 ZG et suivants du code général des impôts. Si l'objectif est d'alourdir la fiscalité applicable à ces opérateurs, il paraît plus pertinent d'agir à ce niveau-là,

nous considérons que la prévention doit passer par un travail de pédagogie et de sensibilisation et que les taxes comportementales ont très souvent atteint les limites de leur efficacité, au vu des niveaux qu'elles affichent déjà. Nous leur préférons des actions plus ciblées. J'aurai l'occasion de

Depuis toujours, l'alcool représente un fléau social et sanitaire. Il continue de détruire des familles et des vies. Son ampleur, loin de décroître, se stabilise.

Le coût de ces séjours hospitaliers est estimé, par le ministère, à 2,64 milliards d'euros- c'est précis -, et les conséquences de la consommation excessive d'alcool restent l'un des tout premiers motifs d'hospitalisation en France. De fait, la France a une position toute particulière, puisqu'elle est le deuxième pays le plus consommateur d'alcool, avec 16 % de la population, en moyenne, consommant du vin de six à sept fois par semaine. Ce danger latent pour la population doit être réduit au maximum, et nous devons tout faire pour que la consommation ne devienne jamais une pratique excessive- c'est bien cette pratique excessive que nous ciblons ici. À cet égard, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la France serait particulièrement concernée par le nombre de cancers évités

il serait peut-être utile, à ce stade, d'attendre les résultats de l'action inscrite dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers, qui vise précisément à réduire les consommations d'alcool à risque.

des jeunes. Les professionnels sociaux et médico-sociaux sont aussi mobilisés pour opérer un repérage précoce des situations de consommation excessive. Pour ces raisons, et même si, sur le fond, je partage l'idée qu'il faut lutter contre la consommation excessive d'alcool,

Mme Raymonde Poncet Monge. Présent dans des milliers de produits alimentaires de consommation courante, l'aspartame est l'édulcorant intense le plus utilisé au monde. Pourtant, dès son apparition dans les années 1960 aux États-Unis,

des sucres par [de l'aspartame] dans les produits au goût sucré ». Ainsi, selon l'agence, l'objectif de réduction des apports en sucre doit être atteint, notamment, par la réduction globale du goût sucré de l'alimentation dès le jeune âge, et non en cherchant à le préserver par le biais d'une substitution. Si l'Agence européenne du médicament a conclu, en 2013, que l'aspartame et ses produits de dégradation étaient sans danger pour la consommation humaine, d'autres études ont depuis lors évoqué ses dangers. Une étude parue en décembre 2018 dans la revue spécialisée dévoile que dévoile que la consommation de boissons contenant de l'aspartame favorise l'obésité et a donc une responsabilité dans l'ensemble des maladies chroniques qui y sont associées. En tout état de cause, nous devons

De ce point de vue, la progressivité est indispensable, car elle permet d'aboutir à terme à une taxation dissuasive, tout en laissant aux industriels, c'est important, le temps de s'adapter. Par ailleurs, nous considérons qu'il est urgent de mener ... Votre temps de parole est écoulé, ma chère

Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les grands industriels de la bière ont pour cible les 18-25 ans, voire les enfants de moins de 18 ans.

-à l'aide d'arômes, de sucres ou d'édulcorants ; un prix compétitif, inférieur à celui des bières artisanales aromatisées ; enfin, un empaquetage conçu pour attirer l'oeil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit « tendance ». Cependant, les jeunes sont plus susceptibles de développer une addiction et, ainsi, de s'exposer tôt à des risques sociaux et sanitaires. Les niveaux de consommation d'alcool dans cette catégorie de la population sont aujourd'hui très préoccupants. De plus en plus de jeunes, d'ailleurs, sont concernés par les risques de coma éthylique. Le cerveau de l'adolescent étant plus vulnérable aux substances psychoactives que le cerveau adulte,

La bière est consommée par les jeunes à 63,5 %. La précocité de l'entrée dans la consommation régulière accroît les risques de dépendance ultérieure, avec tous les dommages à long terme que nous connaissons.

Ainsi, une canette de 50 centilitres d'une bière à 8,5 degrés d'alcool représente trois unités standards d'alcool, alors que la recommandation officielle est de ne pas dépasser deux unités par jour-

Dans une démarche de prévention des risques liés à l'alcoolisation excessive, nous proposons, par cet amendement, d'instaurer une taxation dont l'objectif est double : limiter l'achat et la consommation de ce type de bière

excède 2,8 % en volume, ce droit est doublé, pour atteindre 7,68 euros par degré d'alcool pur par hectolitre. Aussi, plutôt que de créer d'emblée une nouvelle taxe, il serait peut-être préférable de dresser le bilan de la taxe existante,

mais elle relève plutôt- passez-moi l'expression -d'un certain bricolage fiscal. Peut-on vraiment parler d'un financement de la perte d'autonomie, alors qu'il est prévu des quantièmes pour réussir à atteindre péniblement le milliard d'euros ?

L'article 17, qui organise les transferts financiers pour 2022 entre l'État et la sécurité sociale, démontre, me semble-t-il, que nous sommes arrivés au bout d'un système ; le financement de la branche famille par une ponction sur la taxe sur les salaires de l'hôpital en est la preuve. Le remplacement des cotisations sociales par la CSG et les autres taxes atteint un niveau jamais égalé et remet en cause le pilier fondateur de la sécurité sociale,

Comme je l'ai déjà indiqué en défendant notre motion tendant à opposer la question préalable, nous refusons cette fiscalisation et cette étatisation toujours plus fortes de la sécurité sociale et défendons un système fondé sur la cotisation sociale et sa gestion

de masquer finalement le manque d'ambition du Gouvernement en matière de politique familiale, comme l'a d'ailleurs souligné le rapporteur de la commission pour la famille. Il est donc préférable de s'en tenir aux seuls ajustements nécessités par les évolutions de périmètre au sein du régime général, en particulier du fait de la création de la branche autonomie.

que l'excédent de la branche famille qui sera constaté à la fin de l'année soit affecté au financement de la branche maladie pour la prise en charge des indemnités journalières non pas

Le scrutin est clos. le résultat du scrutin. Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence,

Cet amendement vise à rétablir la compensation intégrale par l'État des pertes de recettes pour la sécurité sociale de mesures d'exonération de cotisations sociales. Sur les 67 milliards d'euros d'exonérations et d'allégements de cotisations sociales consentis en 2020, près de 3 milliards d'euros ne sont pas compensés par l'État.

d'autant plus que cette dérogation porte sur les pertes de recettes consécutives, notamment, à l'exonération de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires, à l'exonération de forfait social au titre de l'intéressement dans les petites et moyennes entreprises (PME) et aux réductions du taux de contribution sociale

des débats hier. Enfin, le solde des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour 2022 est amélioré de 1,2 milliard d'euros par rapport au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

ce n'est pas ainsi que l'on va rétablir l'équilibre du système de retraite par répartition. En conséquence, le déficit de la branche retraite s'élèverait à 6,4 milliards d'euros à l'horizon 2025 pour le régime général et même à 9 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes vieillesse,

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

droit. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

pour les aligner sur le régime de remboursement des consultations en présentiel. L'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale prévoit le principe d'une participation restant à la charge de l'assuré après le remboursement par l'assurance maladie de certains actes et consultations. Le respect, ou non, du parcours de soins est naturellement pris en compte. En l'état actuel du droit, le professionnel de santé et le patient doivent être présents au sein du cabinet de ville ou de l'établissement de santé lors de la consultation Je vous propose de modifier cet article pour permettre aux patients d'être situés à distance durant cet acte, seul le médecin devant être présent en ville ou dans l'établissement ou le centre de santé Nous devons mieux réguler les téléconsultations en favorisant le respect des parcours de soins et des bonnes pratiques de la part des opérateurs et en responsabilisant les assurés. Tel est l'objet de cet amendement.

En revanche, à compter du 1 janvier 2022, le remboursement des téléconsultations retombera dans le droit commun du remboursement des actes en télésoin et pourra, à ce titre, faire l'objet d'une participation forfaitaire de l'assuré. Les téléconsultations seront en outre de nouveau soumises à l'exigence du parcours de soins coordonnés.

Ce sous-amendement vise à préciser que l'interopérabilité doit également être sémantique et à intégrer dans le texte la notion de nomenclature. La nomenclature interopérable se trouve au coeur du développement des systèmes d'information de santé.